La séance est reprise.

C'était la victoire d'une équipe métissée, vite surnommée « black-blanc-beur ». Comme le notait le sociologue et ancien ministre Azouz Begag, chacun pouvait alors s'identifier à une histoire à travers un joueur : Zidane pour les personnes originaires d'Afrique du Nord, Karembeu pour les Kanaks, Djorkaeff pour les Arméniens, Henry pour les Antillais, Lizarazu pour les Basques. Rien de tel en 2018 ! Nos champions n'ont qu'une expression à la bouche : « Vive la République, vive la France Ils disent leur fierté d'être Français, chantent la jusque sur le perron de l'Élysée et refusent d'être renvoyés à leurs origines. Ainsi, quand le site Sporf

On ne peut que se féliciter de cette initiative, qui montre que cette équipe multicolore incarne et revendique avec éclat l'unité nationale et les valeurs de la République, à rebours de toute velléité identitaire. Barack Obama ne s'y est d'ailleurs pas trompé lorsqu'il a déclaré : « Regardez l'équipe de France qui vient de

allons-nous tous continuer à faire vivre cette promesse de l'unité nationale que nos compatriotes ont découverte, ou redécouverte, avec ferveur ?

En tout cas, elle n'est pas neutre. C'est parce qu'elle n'est pas neutre qu'elle a suscité autant de réactions : certains dénigrant le caractère de cette équipe, d'autres, au contraire, le

Obama, qui s'est exprimé à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Ce n'était probablement pas neutre dans son esprit, et ce n'est clairement pas neutre dans le mien. Au fond, ce Au fond, ce qui est le plus notable dans cette victoire, c'est ce que les joueurs en disent eux-mêmes. Bien souvent, nous avons la tentation de faire dire aux sportifs, surtout lorsqu'ils sont victorieux, des choses qui nous arrangent.

De toute évidence, cet homme aurait dû être jugé et sanctionné. M. Bruno Roger-Petit, porte-parole de M. Macron, a avancé ce matin une défense curieuse. Il a révélé que M. Benalla n'était pas seul, était accompagné d'un gendarme réserviste, M. Vincent Crase, employé de La République En Marche, selon la presse, et occasionnellement recruté par le service de sécurité de l'Élysée. Quelle était la mission

Sont-ils prêts à venir dans les meilleurs délais ? La commission d'enquête demandée par nos amis du groupe GDR et d'autres groupes à l'Assemblée nationale doit être mise en place pour que la vérité soit établie et pour qu'il soit mis un terme à l'intervention des barbouzes du nouveau monde dans les mouvements sociaux. Cette affaire d'État est grave. Elle symbolise la violence sociale mise en oeuvre par votre gouvernement, sur directive du Président de la République. L'arrogance et le mépris affichés chaque semaine par le nouveau pouvoir mettent en péril l'équilibre social et le pacte républicain. Ces faits ne sont pas anecdotiques. Il ne s'agit pas d'un faux pas. Ils sont l'expression d'une politique autoritaire, dont les excès doivent être dénoncés.

Cette rigueur et cette transparence me conduisent à préciser plusieurs points. Premièrement, il est clair que si l'individu que vous avez mentionné était présent aux côtés des forces de l'ordre le 1 mai, ce n'était en aucun cas dans le cadre d'une mission qui lui aurait été confiée. Il avait été autorisé à titre personnel à assister en tant qu'observateur aux opérations de maintien de l'ordre. Par qui ? Avec un

Ça ... Mesdames, messieurs les sénateurs, vous dites à juste titre qu'il s'agit d'une question sérieuse. J'essaie donc d'y apporter des réponses sérieuses et précises. Je n'ai pas le sentiment de faire le pitre

il est clair qu'un comportement de ce type exigeait une réaction de la part de l'employeur de cet individu.

été mis à pied durant quinze jours, sans traitement, à compter du 4 mai. C'est la raison pour laquelle je dis que la décision a été prise très rapidement. Vous le savez, madame la présidente Assassi, une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de Paris.

parce que c'est naturel de le dire et parce que c'est ce que nous souhaitons. L'affaire est désormais aux mains de la justice.

Que faisait ce collaborateur du Président de la République aux côtés des forces de l'ordre, prétendument comme observateur, et accompagné, nous l'avons appris ce matin, d'un salarié de La République En Marche ? Bonne question ! Qui l'a missionné pour cela ou lui en a donné l'autorisation ? Quelles consignes avaient reçues les policiers par rapport à la présence et aux actes d'Alexandre Benalla ? Plus largement, y a-t-il eu d'autres faits de même nature depuis un an, lors d'autres manifestations ? ? Ah ... Alors que le Premier ministre nous parlait à l'instant de transparence, pourquoi cette affaire, rendue publique hier par la presse, a-t-elle été dissimulée et qui a pris la décision de l'étouffer ? Qui peut accepter que, malgré des faits aussi graves, M. Benalla continue apparemment de travailler à l'Élysée ? Bonne question ! Pourquoi n'y a-t-il pas eu de saisine immédiate du procureur de la République, en application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, ce qui aurait été le minimum en cette affaire ? Absolument, c'est la loi ! Certes, le parquet vient d'ouvrir une enquête préliminaire, mais cela n'aurait pas eu lieu sans les informations du journal. Voilà qui est très grave ! Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons donc la vérité sur cette affaire ... Oui ! ... et, enfin, une réaction à la mesure de sa gravité.

vient nuire à l'image et au professionnalisme de leur action. Les forces de l'ordre se sont en effet attachées, pendant la manifestation du 1 mai,

faits. Je veux souligner que ces deux personnes n'avaient évidemment aucune légitimité pour intervenir. Elles avaient été autorisées par la préfecture de police de Paris à assister en tant qu'observateurs- et observateurs seulement -au déroulement d'un service de maintien de l'ordre d'une manifestation.

Ces manifestations sportives engendreront un certain nombre de chantiers dans toute la région francilienne. C'est ainsi que le département de la Seine-Saint-Denis devrait construire huit piscines supplémentaires. La célèbre gare du Nord devrait tripler de volume et le réseau de transport francilien devrait, quant à lui, connaître de nombreuses ramifications afin de couvrir ces événements, désengorgeant les transports urbains. Pourtant, force est de constater que ces chantiers ne cessent de prendre du retard. À ce rythme, le fameux « chantier du siècle », selon les mots du Premier ministre, ne verra pas le jour aux dates prévues. En effet, les experts ne tablent aujourd'hui sur une opérationnalité du métro automatique du Grand Paris Express qu'à l'horizon de 2030. Ces retards ont malheureusement conduit à des arbitrages, qui font aujourd'hui des victimes dans les territoires les plus périphériques. comment justifier nos ambitions pour l'immense de Paris-Saclay, pôle scientifique et technologique à renommée internationale, qui ne sera desservi qu'en 2025 ? Si ces événements sportifs sont une formidable opportunité, nous devons tout faire pour qu'ils soient une chance économique, sociale et territoriale pour notre pays. C'est pourquoi nous devons nous assurer, avec la plus grande fermeté, que toutes ces constructions et tous ces aménagements du réseau servent le pays dans l'immédiateté de ces événements et dans la construction de l'Île-de-France de demain. Pour toutes ces raisons, madame la ministre, je souhaite savoir quelles mesures vous comptez prendre pour pallier les retards d'extension du réseau en matière de couverture « transport » des territoires ultrapériphériques et quels équilibres vous comptez fixer pour rendre vos arbitrages sur la construction différenciée de certaines lignes. La parole

je vous remercie de votre question. Le Grand Paris Express est un vrai projet d'avenir pour la région capitale. À terme, il va transformer, pour le meilleur, la vie de millions de Franciliens. Ce développement est d'ailleurs d'une ampleur considérable, vous l'avez souligné. Avec 200 kilomètres de lignes nouvelles, 68 nouvelles gares, c'est un défi absolument hors norme, mais nous avançons. Vous le savez, le 22 février dernier, le Premier ministre a confié la réalisation intégrale du schéma d'ensemble d'ensemble et confirmé, après avoir consulté les élus franciliens, que le phasage annoncé était aussi réaliste que crédible. Bien sûr, et vous avez raison de le noter, l'échéance des jeux Olympiques de 2024 est une date clé. toutefois à vous assurer, au nom du Gouvernement, que l'ensemble du projet ne se fera pas au détriment des territoires. Ah ! Je ne crois pas que la ligne 14 qui sera livrée en 2024 et transportera un million de personnes par jour ne concernera que les jeux Olympiques. Les nouvelles lignes de métro participeront avant tout au développement des territoires qu'elles desserviront. Ah oui ? Nous gardons bien à l'esprit que ce projet, qui est d'intérêt national, est actuellement financé intégralement par les Franciliens. Il est donc fait par et pour les Franciliens, et nous nous attelons à trouver des financements complémentaires. Ah bon ? Lesquels ? C'est tout l'objet de la mission qui a été confiée par le Premier ministre à Gilles Carrez. Si ses indications sont justifiées, elles devront être intégrées, et elles Enfin, concernant la question spécifique du rephasage du calendrier, la ministre chargée des transports, Élisabeth Borne, a confié une mission au préfet d'Île-de-France. Avec Île-de-France Mobilités, il devra définir et mettre en oeuvre les offres complémentaires de transport nécessaires.

ce qui placera brutalement les CCI dans le champ concurrentiel, en menaçant leur existence ; nous en reparlerons. Vous en avez aussi profité pour jouer au bonneteau- comme d'habitude -, une nouvelle fois au détriment des collectivités locales. En effet, vous avez annoncé que le désengagement de l'État dans les CCI serait compensé, pour les entreprises, par « une baisse à due concurrence de la CVAE et de la CFE Cela revient, pour le Gouvernement, à faire un triple mauvais coup : réaliser des économies budgétaires en se désengageant des CCI pourtant déjà exsangues ; faire supporter aux collectivités locales la compensation du désengagement de l'État et réaliser à bon compte un allégement de la fiscalité des entreprises punir une nouvelle fois les collectivités locales en leur imposant ce nouveau transfert de charges, qui ampute à la fois leur autonomie fiscale et leur autonomie financière. C'est un très vilain coup, parmi tant d'autres, porté par Bercy, et ce en contradiction avec les annonces du Président de la République lors du Congrès sur le meilleur accompagnement des territoires et les vôtres devant la commission des affaires économiques du Sénat il y a quelques mois. Monsieur le ministre, vous devez maintenant préciser vos funestes projets : au sein des collectivités, qui paierait, comment et à quel rythme ce nouveau désengagement de l'État ?

le Gouvernement a en effet décidé d'engager une réforme ambitieuse des chambres de commerce et d'industrie, dont les principes ont été présentés par Bruno Le Maire, le 10 juillet dernier, à l'ensemble des présidents de CCI réunis en assemblée générale. Ce qui est proposé, c'est de changer d'approche et de logique, de lancer, en lien étroit avec les CCI elles-mêmes, une réforme d'ampleur du réseau pour lui redonner un sens et en refaire un outil de politique publique sur lequel l'État peut s'appuyer. Nous souhaitons que les CCI restent des établissements publics de l'État, présents dans tous les territoires. Cette réforme des CCI, nous allons la faire non pas contre les présidents de CCI ou contre les salariés, mais avec eux. Nous repensons le périmètre des missions financées par la taxe affectée. Il s'agit d'une ressource publique prélevée sur les entreprises, dont nous devons à ce titre justifier l'usage et assurer l'efficience. Nous devons repenser la gouvernance et le pilotage de ce réseau. Trop souvent, les CCI ne savent pas parler d'une seule voix, elles n'offrent pas la même qualité de service aux entreprises sur tout le territoire. Nous souhaitons donner un rôle central de pilote à CCI France, car il ne peut y avoir d'opérateurs de l'État sans un pilotage resserré. Enfin, dans cette réforme, nous accompagnerons accompagnerons le réseau des CCI et, surtout, leurs salariés. Il s'agit ici de repenser le rôle des CCI et leur mode d'organisation, d'accompagner les salariés dans ces évolutions et non de transférer des budgets d'une poche à l'autre. Il s'agit donc bien de trouver au sein des CCI et dans une nouvelle vision stratégique les leviers de leur transformation. Vous

comme votre rapporteur général de l'Assemblée nationale sur d'autres sujets, la grande imprécision relative aux conséquences des décisions fiscales que vous sortez du chapeau. La

Le groupe Union Centriste s'associe pleinement aux félicitations du Sénat adressées à l'équipe de France de football, qui nous a remplis de fierté, de joie et d'enthousiasme, comme des millions de Français qui sont descendus dans les rues pour fêter cet événement dimanche dernier.

Sur le plan matériel, nous aimerions savoir combien de véhicules ont été brûlés, combien de magasins ont été saccagés et quel en est le coût. Quel est le nombre d'arrestations

Vincent Delahaye, tout comme vous, je tiens à saluer l'action des forces de sécurité intérieure, qui ont été pleinement mobilisées pour les festivités des 13 et 14 juillet,

où la menace était particulièrement importante. Lorsque vous êtes ministre de l'intérieur et que vous organisez de telles manifestations,

nous a permis d'assurer des périmètres de protection, sans lesquels il aurait été impossible d'organiser ces grandes manifestations. Nous avons mobilisé le maximum d'hommes et de femmes : 110 000 policiers et gendarmes, 44 000 sapeurs-pompiers, militaires et volontaires, l'ensemble des associations agréées de sécurité civile. C'est vrai, vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, après ce match, après que celles et ceux qui soutenaient l'équipe de France sont partis, il est resté dans quelques villes

Les individus ont été mis en garde à vue. La qualité de ces interpellations et des investigations réalisées par les fonctionnaires de police a été telle que des réponses pénales immédiates avec un certain nombre d'incarcérations. Nous sommes en train de regarder les images vidéo et des suites seront données à chaque action contre l'ordre public.

Catherine Morin-Desailly, a organisé ici même un grand colloque intitulé « Comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique ? ». Ce fut un moment très intéressant, notamment grâce à l'intervention de grands responsables de l'audiovisuel public

pour la réforme de l'audiovisuel public en France et nous indiquer le cadre global dans lequel le Gouvernement entend inscrire ce grand chantier ? La parole

Vous le savez, aujourd'hui, on ne peut plus envisager la télévision de la même manière avec Netflix, avec YouTube et avec un jeune public qui regarde de plus en plus les images sur son smartphone plutôt que sur le poste de télévision familial. Notre conviction, qui a été confirmée par la commission de concertation, c'est que le service public audiovisuel est une nécessité et une force, à condition qu'on l'aide à se transformer et que l'on ait une véritable stratégie, au-delà de tout conservatisme. les sociétés de l'audiovisuel public doivent passer d'une logique de diffuseur à une logique d'éditeur de contenu avec quatre grandes priorités. La première, c'est le renforcement de l'offre de proximité, que j'ai déjà détaillée, avec un triplement des programmes de France 3, des coopérations beaucoup plus étroites avec France Bleu et des expérimentations qui démarreront dès la rentrée pour s'adapter à chaque territoire et partir de ces territoires. La deuxième priorité, c'est l'enrichissement et l'évolution de l'offre de programmes pour les jeunes, ce qui est confirmé par la commission de concertation. Cela implique de maintenir une très forte ambition dans le domaine des programmes pour la jeunesse, en particulier dans l'animation, qui est une filière d'excellence, et de proposer des contenus éducatifs

Il s'agit de sortir les outre-mer de la périphérie pour leur garantir une véritable présence dans la programmation de toutes les chaînes de France Télévisions. Cette juste représentation sera accompagnée d'engagements précis dans le cahier des charges, qui donneront lieu à un groupe de travail associant les parlementaires concernés et les sociétés.

qui joueront un rôle de tête de réseau dans le groupe. Nous enrichirons également l'offre numérique, et les outre-mer passeront en haute définition, ce qui permettra, à l'échéance de 2020, de libérer le canal hertzien de France Ô, tout en augmentant la visibilité des outre-mer. Le défi numérique nécessite un renforcement des investissements des sociétés dans le numérique, qui permettra de bâtir une stratégie fondée sur l'excellence technologique, sur une ergonomie souple et fluide, sur une expérience utilisateur de grande qualité et sur des environnements qui sécurisent ... Il faut conclure, madame la ministre

La société MSC, deuxième transporteur mondial de conteneurs, vient d'annoncer sa décision de quitter le port de Bordeaux, en raison de l'incapacité de ce dernier à remettre en service le terminal du Verdon une mauvaise nouvelle de plus pour ce grand port maritime, pris dans une spirale négative depuis plusieurs années de mauvaise administration. Cette annonce signifie une diminution de 50 % du trafic de conteneurs et des dizaines d'emplois directs ou indirects condamnés. J'ai une pensée particulière pour les pilotes de la Gironde, dont je suis la marraine d'un bateau et qui sont face à des choix cruciaux de sécurité. La ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine sont mobilisés pour tenter de sauver une activité portuaire qui fait sens dans l'ouverture de la France au monde par sa façade atlantique. Depuis la réforme portuaire de 2008, les grands ports maritimes restent les derniers à conserver le statut d'établissement public sous responsabilité de l'État. Cependant, il manque à ces ports, tout du moins au port de Bordeaux, une vision stratégique territorialisée. Ce port est éclaté sur sept sites différents, dont une partie en estuaire. Il ne peut être géré comme n'importe quel autre grand port de France. La région Nouvelle-Aquitaine apparaît donc comme la seule et unique échelle capable de prendre en compte ses spécificités, en complémentarité avec le port régional de Bayonne et en synergie avec celui de La Rochelle. En transférant cette compétence à la région, l'État permettrait de faire émerger un projet qui fédérerait les acteurs et ne les diviserait plus comme aujourd'hui. L'État y resterait néanmoins un acteur central pour l'accomplissement de ses missions régaliennes liées à la sécurité maritime, au contrôle des flux, ainsi que pour sa compétence en matière de dragage de l'estuaire. Madame la ministre, nombre d'élus et d'acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine attendent la régionalisation de ce port. Cette question stratégique sera-t-elle abordée dans votre projet de loi d'orientation sur les mobilités ? Vous héritez d'une situation complexe. Malheureusement, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Il vous faut agir vite !

est, pour le Gouvernement, un enjeu majeur. Vous savez d'ailleurs que, le 21 novembre dernier, à l'occasion des Assises de l'économie de la mer, le Premier ministre a réaffirmé son engagement en faveur du développement, de la compétitivité et de l'attractivité des ports français. Nous souhaitons

et réformé. Pour ce faire, nous nous concentrons non seulement sur la transformation du modèle économique des ports, mais aussi sur la recherche d'une meilleure complémentarité entre l'ensemble des ports français, ce qui exige la mise en place d'une nouvelle gouvernance. gouvernance. Le Gouvernement souhaite que cette gouvernance soit mieux partagée avec les collectivités qui comptent des grands ports maritimes à vocation plutôt nationale, en particulier ceux de la façade atlantique. raison pour laquelle nous avons chargé le préfet de Nouvelle-Aquitaine d'une mission de concertation auprès de toutes les parties prenantes, qui complétera un audit financier en cours. L'option de la décentralisation du port de Bordeaux est, elle aussi, en discussion. Les résultats de cette concertation seront donc déterminants pour nos échanges à venir. assurée, madame la sénatrice, que, au-delà de la gouvernance, la préoccupation du Gouvernement est de redonner au port de Bordeaux des perspectives stratégiques de développement et de lui donner les capacités de les mettre en oeuvre. La parole

pour le groupe socialiste et républicain. Ma question s'adresse à Mme la ministre des sports. Les festivités saluant le fantastique parcours sportif de l'équipe de France de football sont encore dans tous les esprits, et les échos de ce moment de ferveur populaire et de communion nationale résonnent toujours. Comment capitaliser sur ce formidable événement, au moment où les débats se poursuivent sur la gouvernance du sport et alors qu'approche le débat budgétaire pour l'année prochaine ? Nous souhaitons mettre en perspective cette belle aventure populaire, source de joie et d'inspiration, avec les interrogations que suscite la politique sportive du Gouvernement. Le 9 juillet dernier, devant le Congrès, le Président de la République a présenté sa vision politique sur de très nombreux sujets. Force fut de constater un absent : le sport. De même, les moyens budgétaires mobilisés dans la loi de finances pour 2018 au bénéfice de cette politique publique ont connu une régression. joueurs de l'équipe nationale présentent vingt-trois parcours de formation de très grande qualité, bien souvent dans des clubs aux moyens modestes. Il importe de préserver cette richesse associative. Or ces clubs traversent une période difficile, caractérisée par la baisse des dotations des collectivités, la réduction du nombre de contrats aidés, l'ubérisation du sport, le manque de reconnaissance pour le bénévolat, ainsi que la diminution en 2018 des crédits du Centre face à l'afflux probable de nouveaux licenciés à la suite de l'engouement provoqué par cette victoire, comment allez-vous favoriser l'accueil de tous ces jeunes, et pas seulement dans le football ? Plus largement, le moment n'est-il pas venu de proposer un projet de loi de programmation budgétaire pour le sport, afin de préparer les jeux Olympiques de 2024 à Paris dans les meilleures dispositions, animé par des ambitions fortes dans la construction de l'héritage olympique, par-delà la recherche de médailles, avec l'augmentation du nombre de pratiquants, le développement des équipements de proximité, le désengorgement de la filière des métiers du sport ou bien encore la promotion du sport scolaire ? Comment entendez-vous relever ces défis ?

? Il y a encore une heure, je présidais le dernier comité de pilotage de ce chantier. Tous les acteurs étaient présents. collectivités territoriales, des mouvements sportifs et du monde économique ont salué la très grande qualité de ce travail collectif et ils ont jugé historique le résultat auquel nous étions parvenus. Historique, car, depuis le 13 septembre dernier, le sport français est au rendez-vous avec l'histoire, et c'est le genre de rendez-vous qu'on n'a pas le droit de manquer. Cette nouvelle gouvernance va conduire à une mutation économique du modèle sportif français, ... Avec une baisse ce n'est pas le rôle de l'État de financer durablement les clubs. L'État accompagnera les acteurs associatifs dans cette période de transition- c'est pourquoi j'ai décidé de libérer une enveloppe de 5,6 millions d'euros pour le soutien aux clubs en difficulté mais le changement doit avoir lieu vers un modèle économique moins dépendant des fonds publics. C'est cela l'autonomie du mouvement sportif. Pour le reste, vous le savez comme moi, la discussion budgétaire est en cours. Nous devrons trouver les moyens de financer nos ambitions en matière de haute performance et d'accès à la pratique, car le sport ne peut avancer que sur deux jambes. La

Monsieur le Premier ministre, vous êtes ici devant la représentation nationale, devant des élus de la Nation. La Constitution nous confie deux missions : faire la loi et contrôler l'action du Gouvernement. Nous avons le sentiment que, depuis quelque temps, notre tâche n'est pas simplifiée. Concernant la fabrique de la loi, après un premier trimestre législatif peu dense au cours duquel le Gouvernement n'a présenté aucun texte important, nous faisons face à un embouteillage- et je n'évoque même pas les commissions

Nous ne comptons plus les amendements du Gouvernement qui modifient substantiellement les projets de loi la nuit précédant le débat. Nous avons atteint l'apothéose avec l'amendement annoncé par le Président de la République, qui a balayé d'un revers de main le volet « chômage » du projet de Monsieur le Premier ministre, la totalité des informations dont nous avons besoin pour légiférer ou contrôler ne nous parvient pas toujours exhaustivement dans un délai raisonnable. Nous avons besoin de plus de transparence de la part du Gouvernement. Qu'est devenu le schéma d'emplois 2019, usuellement annexé aux documents de préparation du débat d'orientation budgétaire ? Nous aimerions connaître vos projets et vos objectifs en matière d'emplois publics, ministère par ministère. Pouvez-vous nous expliquer par quelle logique la presse dispose du rapport du Comité Action publique 2022, alors que notre collègue Christine Lavarde, membre de cette instance, n'en a même pas eu connaissance ? pas eu connaissance ? Le Parlement mérite d'être respecté et personne, pas même le Président de la République, ne peut prétendre incarner à lui seul l'édifice républicain. Comment comptez-vous corriger ce qui pourrait être interprété comme de la défiance et du mépris vis-à-vis du Parlement ?

la façon dont nous envisageons la transformation de l'action publique ou encore l'utilisation d'un travail d'experts qui nous a été rendu. Je vais essayer de répondre, sinon à toutes ces questions, du moins de la façon la plus claire possible.

que sur un travail d'experts qui nous a été rendu pour nourrir notre réflexion. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, monsieur le sénateur, malgré un certain brouhaha ... Le Gouvernement n'est

Dans un entretien accordé à un quotidien national, vous avez écarté l'idée de toucher au taux réduit de TVA dans la restauration, estimant « que l'augmentation des impôts n'était pas la bonne solution ». Vous semblez toutefois valider en creux l'idée d'un abandon des taux réduits applicables à la rénovation énergétique et à l'amélioration du bâti. À l'heure où les travaux de rénovation stagnent et où l'État souhaite lutter contre la précarité énergétique, la suppression de ces taux réduits pénaliserait les ménages les plus modestes et produirait des effets désastreux pour le secteur du bâtiment. Les travaux de rénovation représentent près de 60 % des 135 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel du secteur du bâtiment, notamment grâce au taux réduit de TVA, dont vous ne pouvez ignorer l'effet sur l'activité économique de notre pays. Un relèvement du taux de TVA, donc des prix, entraînera une baisse du volume des travaux déclarés, c'est-à-dire une hausse du travail au noir, et, par conséquent, la destruction de milliers d'emplois.

comme l'a bien exposé le Premier ministre, tous les ministères sont actuellement engagés, chacun dans leur champ de compétences, dans une démarche vertueuse d'évaluation de leurs missions et des dispositifs fiscaux et non fiscaux qui les concernent, afin d'identifier les réformes nécessaires à une plus grande efficacité. C'est tout le sens du programme Action publique 2022, lancé en février dernier. Dans ce cadre, le ministère de l'économie et des finances mène une revue des aides budgétaires et fiscales aux entreprises, afin d'évaluer leur efficience économique au regard du coût qu'elles représentent pour les finances publiques. Ces aides font également l'objet de nombreuses concertations avec les associations et fédérations d'entreprises. Cela ne signifie pas qu'elles ont vocation à terme à être remises en cause. Le ministre de l'économie et des finances a par ailleurs annoncé lors de la commission d'évaluation des politiques publiques qu'il souhaitait associer les parlementaires à cette démarche d'évaluation. Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance pour les secteurs concernés des taux réduits de TVA, qu'il s'agisse du taux de 10 % ou de celui de 5,5 % dont bénéficient les travaux de rénovation. La ligne du Gouvernement reste la même : rechercher un impact optimal pour ces réformes en faveur de l'activité économique et de l'emploi. Ce sont donc les dispositifs les moins efficaces à cet égard qu'il faut modifier ou supprimer. Lors du congrès national de la Fédération française du bâtiment, Bruno Le Maire a rappelé l'attention particulière qu'il portait au bâtiment, en annonçant notamment des évolutions positives pour ce secteur : le relèvement de 5 % à 20 % des avances sur les marchés de travaux passés par l'État pour les PME

en train de frapper un manifestant à terre alors que ce dernier avait été isolé par les CRS. Cela s'est passé le 1 mai dernier, et celui qui était alors chef de cabinet adjoint du Président de la République arborait un casque des forces de l'ordre. Son parcours n'est pas exempt d'incidents. Arnaud Montebourg, qui l'avait recruté comme chauffeur, s'en était séparé au bout d'une semaine, il avait provoqué un accident de voiture et voulait prendre la fuite. Il y a plus d'un an, il a arraché l'accréditation d'un journaliste de la rédaction de avant de l'évacuer d'un meeting de M. le Président de la République. Ce qui s'est passé le 1 mai n'a échappé ni au Président en a été informé, ni à son directeur de cabinet. Une sanction est tombée discrètement, aussi dérisoire que symbolique. Madame la garde des sceaux, pourquoi avoir attendu que les faits soient rendus publics pour que la justice se saisisse et ouvre une enquête préliminaire ? Pouvez-vous nous donner la raison pour laquelle le cabinet du Président de la République n'a pas, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, saisi lui-même le procureur de la République ?

loi constitutionnelle. Je crois en un ordre républicain. Seules les forces de sécurité intérieure sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre.

les forces de l'ordre ont assuré avec calme le droit à manifester d'un certain nombre de personnes.

on pense être au-dessus des lois ! Eh oui ! Absolument ! Quelles que soient les suites de cette affaire affligeante, l'Élysée, en ayant tenté d'étouffer les faits et en ne saisissant pas la justice dès le premier jour, aura failli à son devoir d'exemplarité.

Depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années, les violences antisémites et les provocations islamistes se multiplient dans notre pays. L'imam de Toulouse a récemment tenu des propos que l'on aimerait ne plus jamais entendre sur notre sol. Il a lancé un appel au meurtre des juifs au nom de l'islam et au nom « du respect des commandements divins ». Cet imam est coutumier du prêche haineux et violent. Ses références sont celles des islamistes. Son modèle est celui des Frères musulmans. Il affiche tranquillement son hostilité à la démocratie et sa haine de la France. Il brandit régulièrement la victimisation des musulmans, fustige la loi française et ses choix démocratiques sur fond de réquisitoire contre l'Occident et ses valeurs. Face à cette situation, le maire de Toulouse a procédé à un signalement à la justice, ce qui a fait réagir le parquet, qui a demandé une enquête. En revanche, on ne vous a guère entendu sur cette affaire, monsieur le ministre d'État. J'ai bien cherché, mais

Marseille. L'émotion dans cette assemblée était très forte, et j'y ai condamné avec la plus grande fermeté des propos qui incitent effectivement à la haine. Les actes antisémites se sont multipliés en France ces dernières années et l'on déplore une succession de personnes sauvagement assassinées.

La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Ce quota de 30 % est, à notre avis, largement insuffisant et constituerait une grave et brutale régression sociale pour les droits des personnes en situation de handicap, même si c'est déjà mieux que le taux de 10 %

soit seulement 40 % de la production de logements nouveaux qui, eux-mêmes, ne représentent que 1 % du parc immobilier français. Par ailleurs, les besoins quantitatifs et qualitatifs des personnes handicapées et des personnes âgées en matière de logements ne sont d'ores et déjà pas satisfaits, même avec le quota actuel ce qui tient en partie au fait que les obligations en matière d'accessibilité ne portent que sur les logements neufs. Lesdites obligations ne constituent qu'une chimère, peu respectée du fait des nombreuses dérogations délivrées aux constructeurs concernés.

d'« évolutivité », qui concernerait les 70 % de logements restants, est à notre avis un peu flou. Tout d'abord, comme l'a reconnu le directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers lui-même,

Ce seuil représente, à nos yeux, le minimum acceptable. En outre, ce taux est assorti d'une clause pour ventiler ces logements, afin que chaque étage compte au moins un logement accessible. Je le répète, ce débat est surréaliste, la proposition du Gouvernement inacceptable.

Si le Sénat a heureusement rehaussé le seuil en commission en le fixant à 30 %, ce taux nous semble toujours largement insuffisant. Il y va de la liberté d'installation des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il y va également de leur sociabilité ou, plus prosaïquement, de leur capacité à se rendre dans leur famille ou chez leurs amis. On nous rétorquera que le logement reste évolutif, c'est-à-dire accessible après la réalisation de travaux simples. Or cette notion est tout à fait critiquable, car complètement floue. Enfin, puisque c'est

à côté du local à poubelles ou du local à vélos, réduisant encore la liberté de choix des personnes handicapées. Quel

Xavier Iacovelli, pour explication de vote. « Notre conviction, c'est qu'il faut avancer, non seulement pour les personnes handicapées, mais avec elles, comme membres à part entière et égale de notre société. C'est l'honneur de la France que de promouvoir ainsi une société plus inclusive, fraternelle et solidaire. À peine un an après ces propos tenus par Emmanuel Macron, le Gouvernement présente un projet de loi qui marque un recul sans précédent de notre société pour toutes les personnes en situation de handicap. Pour ce qui est des chiffres, la mission est remplie. Nous discutons depuis des mois pour savoir quel sera le bon taux de logements accessibles à l'avenir 10 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 % ..., on en restera à un taux de 30 % au Sénat. Monsieur le ministre Mézard, dans votre intervention liminaire, lundi dernier, vous avez indiqué qu'il faudrait trouver le point d'équilibre.

brutal pour tous les Français qui aspirent à une société plus ouverte et plus solidaire, brutal pour toutes les associations, pour toutes les personnes handicapées, qui tentent depuis des mois d'infléchir votre décision. Le Président de la République disait vouloir avancer pour les personnes

Avec seulement 6 % de logements accessibles en France, votre mesure va à l'encontre de la nécessité de prendre en compte tant le handicap que le vieillissement de la population et revient sur l'engagement du Président de la République de faire du handicap une priorité du quinquennat. Monsieur le ministre, il est encore temps, à défaut de retirer l'article 18 de votre projet de loi, de retirer au moins votre amendement

D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, je vous invite à aller ce week-end dans un magasin de bricolage, où on trouve tout ce qu'il faut, pour changer votre baignoire en douche à l'italienne. Sauf à mettre la bonde chez le voisin du dessous, je ne sais pas comment vous ferez

l'éclairage se déclenche à distance, avec une télécommande ou sur le mini-ordinateur embarqué sur la chaise roulante. L'éclairage peut même suivre la personne handicapée dans ses déplacements à travers l'appartement ou la maison.

S'il vous plaît, qu'il a vécues dans des moments qui n'étaient pas toujours simples. D'ailleurs, la suite l'a prouvé. Oh ! J'ai l'habitude de prendre mes responsabilités et de les assumer.

% soit utilisé de manière efficiente, dans l'intérêt de la construction et du logement. Les accords que nous venons de conclure avec Action Logement permettront, justement, une meilleure

Cet amendement vise à assurer un taux d'accessibilité de 100 % des parties communes des bâtiments d'habitation collectifs neufs en équipant chaque niveau de ces bâtiments de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Il s'agit ainsi de favoriser l'inclusion sociale des personnes porteuses d'un handicap et de faciliter la conversion des logements adaptables en logements accessibles. Quel

y compris évolutifs, auront un séjour accessible, ce qui suppose des parties communes accessibles. Il est également précisé que tous les logements, y compris évolutifs,

Si l'on considère que des travaux simples, c'est casser une cloison, élargir un couloir, agrandir le tour d'une porte pour pouvoir laisser passer une personne à mobilité réduite

les alimentations en fluides, quels qu'ils soient, et les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes ; ils ne doivent pas impliquer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation en eau, d'alimentation en gaz

L'amendement n° 881 vise à préciser que les bailleurs sociaux devront prendre à leur charge les travaux de mise en accessibilité, sans préjudice des aides fiscales. L'article 1391 C du code général des impôts

? Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur la faisabilité d'un tel répertoire. Quel est l'avis du Gouvernement Monsieur le ministre,

en toiture des bâtiments commerciaux neufs de plus de 1 000 mètres carrés. Il s'agit d'accroître les capacités d'énergie renouvelable en mobilisant les surfaces artificialisées et de favoriser la biodiversité en milieu urbain et périurbain.

nous proposons que cette obligation porte sur une part significative de la toiture et qu'elle soit étendue aux ombrières protégeant les aires de stationnement. L'amendement vise à définir une surface minimale d'au moins 30 % pour améliorer l'opérabilité de cette mesure. Il est désespérant de constater le retard de certaines filières économiques qui ont pourtant tout à gagner avec des dispositifs comme celui-ci. Quand on voit, près des aéroports, des zones commerciales sans un seul panneau photovoltaïque- alors que, compte tenu de leur surface, elles doivent viser l'autonomie énergétique -et sans toiture végétalisée permettant de réduire la chaleur et de faire des économies d'air conditionné, c'est à n'y rien comprendre. Ces zones devraient montrer l'exemple de cette mutation, car elles seraient les premières à bénéficier de la transition énergétique. Pourtant, ce sont elles qui freinent des quatre fers. Mes chers collègues, nous devons faire preuve ici non pas d'idéologie justement, mais de pragmatisme, car nous voyons bien que, sur le terrain, rien ou trop peu de choses se passent. Quel

inventer, par loi d'habilitation, une réglementation thermique des constructions. Il s'agit là d'un amendement de bon sens. Il semble que la reconnaissance de la notion de préfabrication n'entraîne en rien une exonération des normes applicables en matière de construction pour ce type de procédé, y compris de celles qui sont en vigueur outre-mer. Toutefois, la commission a souhaité demander l'avis du Gouvernement afin d'obtenir confirmation sur ce point.

amendement, tel qu'il est rédigé, n'apporte pas de précision supplémentaire, puisque toute construction, préfabriquée ou non, doit se soumettre à la réglementation en vigueur, y compris celle qui est spécifique aux territoires ultramarins.

En effet, alors qu'un consensus semble émerger pour favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'exigence du développement durable, que l'urgence d'une transition énergétique écologique est actée par tous, un projet de loi sur le logement ne peut faire l'impasse sur la question des matériaux de construction. Le secteur du bâtiment est l'un des secteurs les plus émissifs de gaz à effet de serre. De plus, l'utilisation du béton, au fort impact environnemental, n'est pas neutre, notamment parce que sa fabrication demande l'importation de beaucoup de sable. Aujourd'hui, des alternatives existent. Elles sont le plus souvent préconisées par les architectes qui, au-delà des plans de construction, formulent des indications sur les matériaux utilisés. Je pense au chanvre, par exemple, ou alors à l'utilisation de briquettes, fabriquées dans le Nord et utilisées pour la construction. Je pense encore à certains matériaux capables de retenir les gaz à effet de serre : autant d'atouts à valoriser. Outre les vertus écologiques de certains matériaux, un tel processus permet de relocaliser de l'emploi dans certaines zones désertées, de promouvoir des circuits courts et de contrecarrer l'importation de sable venu de loin. Nous souhaitons donc qu'un rapport recense l'ensemble de ces expériences et préconise les évolutions législatives pour favoriser l'utilisation de tels matériaux et le développement de circuits courts. Quel le ministre

n° 418 rectifié. L'article 19 A ajoute un point III à l'article L. 243-1-1 du code des assurances et précise le champ des dommages aux existants couverts par l'assurance décennale obligatoire. Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait d'aligner le champ de l'obligation d'assurance et celui des dommages couverts, en simplifiant la rédaction de cet article. Une rédaction du point II qui engloberait ces deux éléments permettrait également d'éviter une réécriture des clauses types figurant aux annexes I, II et III de l'article A243-1 du code des assurances.

Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait d'aligner le champ de l'obligation d'assurance et celui des dommages couverts, en simplifiant la rédaction de l'article L. 243-1-1 du code des assurances. Une rédaction du point II qui engloberait ces deux éléments permettrait également d'éviter une réécriture des clauses types figurant aux annexes I, II et III de l'article A243-1 du code des assurances.

Il s'agit d'une réponse à une jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a pris le contre-pied de la volonté du législateur lors de l'adoption de l'article L. 243-1-1, point II, du code des assurances, qui définit le champ de l'obligation d'assurance en cas de travaux sur existant. Or opérer cette clarification revient à créer une distinction qui ne se justifie pas entre, d'une part, le champ de l'obligation d'assurance visé par le point II de l'article L. 243-1-1 et, d'autre part, celui des dommages couverts visé par le point Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait d'aligner le champ de l'obligation d'assurance et celui des dommages couverts, en simplifiant la rédaction de l'article L. 243-1-1 du code des assurances et en englobant ces deux éléments.

satisfait : d'une part, l'article 5 de la loi de 1977 n'établit aucune distinction selon le type de construction ; d'autre part, le simple fait de définir la préfabrication n'a pas pour conséquence de l'exonérer de l'ensemble des règles qui sont applicables aux constructions.

L'article 19 crée l'obligation pour le propriétaire d'un terrain constructible de fournir au moment de la vente ou préalablement à la construction d'un nouvel immeuble une étude géotechnique dans les zones exposées au risque du retrait-gonflement des sols argileux. Il renchérit le coût des cessions de terrain sans pour autant que le projet, qui n'est pas nécessairement défini, mobilise en aval les résultats de cette étude géotechnique sommaire. Cette nouvelle obligation pèsera particulièrement sur les fonciers peu chers, en zone rurale essentiellement. Il conviendrait mieux

de rendre obligatoire cette mention sur le certificat d'urbanisme

Il généralise le recours aux procédures de conception-réalisation pour la production de logements sociaux par les organismes d'HLM. Nous avons toujours considéré que le recours à la conception-réalisation ne trouvait de justification que dans son caractère exceptionnel, d'ailleurs strictement rappelé par la loi.

Cette manière de procéder place les architectes sous la dépendance des grands groupes du secteur du BTP, qui n'ont pas nécessairement les mêmes attentes en matière de qualité architecturale du bâti ou de son intégration dans un environnement. Une telle conception représente une rupture avec la déclaration de Davos signée cette année par une vingtaine de pays européens, mais non, il est vrai, par la France, et indiquant que l'objectif de la culture du bâti de qualité est d'atteindre et de maintenir un haut niveau de qualité de l'environnement bâti. Cela passe notamment par le concours d'architectes. Cette qualité, selon cette déclaration, engendre des plus-values sociales essentielles telles que l'amélioration de la qualité de vie, du bien-être, de la cohésion et de l'intégration sociales.

Nous prônons le respect de l'allotissement, qui est une manière de mieux maîtriser les coûts et de développer les filières locales. Nous ne sommes pas, vous l'aurez compris, favorables à la pérennisation de la possibilité, pour les organismes d'HLM, de recourir à ce type de procédure qui, sous couvert de faire vite, se fonde sur une vision purement comptable et commerciale. La

d'un secteur bien particulier, sans aucune évaluation ni justification précise. La loi MOP, qui repose sur le triptyque maître d'ouvrage-maître d'oeuvre-entrepreneur, prévoit, à son article 18, une exception dite de « conception-réalisation », permettant à un même opérateur de remplir ces deux missions. Pour autant, afin d'éviter tout excès, et surtout de maintenir un équilibre entre les différents acteurs économiques, le recours à ce type de marché est strictement encadré, seules deux raisons pouvant le motiver. Depuis 2009, le champ de cette dérogation est encore plus vaste pour les bailleurs sociaux, qui sont exemptés de toute justification de recours aux contrats de conception-réalisation. Cette expérimentation a déjà été prolongée

bilan de l'expérimentation. À ce titre, rappelons que la dernière analyse du dispositif remonte au rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui date de 2013. Autrement dit, nous, législateurs, pourrions graver dans la loi une procédure insuffisamment expertisée, aux conséquences incertaines et potentiellement lourdes, que ce soit en termes de qualité de construction, de coût global, de valeur d'usage pour les habitants ou d'équilibre économique pour l'ensemble du secteur. D'ailleurs, dans son avis, le Conseil d'État soulignait à juste titre que, dans l'éventualité d'une pérennisation de la conception-réalisation, il serait nécessaire « de prendre en compte tant les impératifs auxquels la loi MOP entend répondre que les enjeux auxquels sont confrontés les offices publics de l'habitat ».

Cette mesure représente une atteinte inacceptable au principe de liberté d'accès à la commande publique, consacré par l'article 1 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. L'essence même de ce principe est d'assurer non seulement l'efficacité de la commande publique, mais aussi la bonne utilisation des deniers publics.

20 vise à étendre le recours à la conception-réalisation aux constructions neuves, puisqu'il serait désormais possible lorsqu'un engagement contractuel sur un niveau de performance énergétique rend nécessaire d'associer l'entreprise au stade de la conception. de recourir à la procédure pour toutes les constructions neuves, au motif du simple respect, par exemple, de la réglementation thermique en vigueur, ce qui ferait de la conception-réalisation à une procédure de droit commun pour la réalisation de tous types de bâtiments publics, quel que soit le maître d'ouvrage. Cette généralisation, contraire au principe de l'allotissement et aux règles issues des directives européennes

ce dont notre groupe se félicite, ayant toujours contesté l'utilisation de cette procédure qui place les architectes sous l'autorité des groupes du BTP et rompt avec un principe fort de la loi MOP : la séparation entre la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage.

La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction du maître d'oeuvre de celle de l'entrepreneur chargé de la réalisation de l'ouvrage, étant prévue, à l'article 18, pour les contrats globaux de conception-réalisation. Par ces contrats, le maître d'ouvrage peut confier à un groupement d'opérateurs économiques privés à la fois la conception du projet, l'établissement des études et l'exécution des travaux, soit pour un motif d'ordre technique, soit eu égard à un engagement contractuel d'amélioration de l'efficacité énergétique. Jusqu'au 31 décembre 2018, le II de l'article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics autorise les bailleurs sociaux à utiliser cette procédure sans avoir à en justifier. L'alinéa 1 de l'article 20 du présent projet de loi tend à inscrire cette procédure dans le droit commun de la réalisation de logements sociaux, ce qui paraît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont la décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008 2008 précise, au sujet du contrat de partenariat, « que la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics

à nous parlementaires, de décider en connaissance de cause, notamment au regard des conséquences que cette dérogation peut entraîner pour l'accès des TPE et des PME aux marchés publics. du présent amendement, il est proposé de s'en tenir à la prorogation du dispositif pour une durée de trois ans, conformément à ce que prévoyait le projet de loi initial. Cela nous permettra, ultérieurement, d'évaluer le rapport risques-avantages de cette mesure et ses effets réels sur l'accélération de la construction de logements sociaux. en outre la suppression de l'extension de la dérogation aux CROUS, adoptée en commission.

du bâtiment aux marchés publics. Il ne serait pas satisfaisant que ces entreprises ne soient au mieux que sous-traitantes, de surcroît dans des conditions économiques très souvent en leur défaveur. Il faut donc conforter la liberté d'accès à la commande publique. Cet amendement

présenter l'amendement n° 262 rectifié. La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction du maître d'oeuvre de celle de l'entrepreneur chargé de la réalisation de l'ouvrage. Cette distinction garantit contre tout risque de situation de conflit d'intérêts pour le maître d'oeuvre, puisqu'il ne peut être lié contractuellement avec l'opérateur économique qui réalise les travaux. Toutefois, l'article 18 de la loi MOP met en place une dérogation permet au maître d'ouvrage de confier à un groupement d'opérateurs économiques privés à la fois l'établissement des études- la conception -et l'exécution des travaux- la réalisation. Cette dérogation est encadrée : seuls deux motifs la rendent possible. Jusqu'au 31 décembre 2018, l'article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics autorise les bailleurs sociaux à utiliser cette procédure sans avoir à en justifier. Cette Cette généralisation est contraire aux principes posés par le Conseil constitutionnel Elle est également contraire au principe de l'allotissement et aux règles européennes visant à favoriser l'accès aux marchés des PME et des artisans, puisqu'elle va restreindre de manière significative l'accès à la commande publique des PME, des TPE et des artisans, qui ne pourront plus obtenir de commandes directes dans le secteur du logement social. Une solution de compromis consisterait à maintenir la prolongation de cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2021, pour les seuls bailleurs sociaux, en l'assortissant de l'obligation de réaliser

conduire le projet avec des maîtres d'oeuvre, avec des maîtres d'ouvrage et avec des entreprises de taille diverse -certes, pas nécessairement des TPE,

dit, la question fondamentale ici posée est celle de la liberté et de l'égalité dans l'accès aux marchés publics.

L'application du droit de la commande publique, tout comme la loi MOP, dépend de la nature juridique de l'acheteur. En ce sens, il y a aujourd'hui des différences selon la nature de l'organisme d'HLM qui construit les ouvrages. Les filiales des offices publics d'HLM sont des sociétés de droit privé, privé, qui ne peuvent être créées et financées qu'à l'aide de fonds extérieurs à l'activité du service d'intérêt économique général du logement social. Elles ne bénéficient donc d'aucune aide publique. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de les soumettre à des règles de marché public, au risque d'introduire une distorsion de concurrence par rapport aux autres sociétés de droit privé.

d'aucune aide publique. Juridiquement, elles sont hors du champ du droit des marchés publics. Il n'y a donc strictement aucune raison de les soumettre à des règles de marché public, au risque d'introduire une distorsion de concurrence, comme Mme la

Concernant le volet de simplification, les mesures visant à renforcer la maîtrise d'ouvrage sociale pour maintenir la production ont engendré de vives réactions émanant de l'Ordre des architectes. Il nous paraît essentiel de mettre fin à ces contrevérités. L'assouplissement des règles est présenté à tort comme un risque en matière de qualité architecturale et de transparence de la maîtrise d'ouvrage. Or il n'en est rien. Nous sommes et restons très attachés aux règles de la commande publique et à la qualité des logements que nous construisons, puis gérons sur le long terme. Ces mesures constituent bien au contraire un moyen de redonner aux organismes d'HLM la possibilité d'adapter, en toute responsabilité, le choix de procédure au contexte et aux besoins d'un projet et de rester ainsi une référence en matière d'innovation, de durabilité, d'adaptabilité et de qualité d'usage. Ne nous trompons pas de débat : l'important aujourd'hui est de pouvoir répondre aux impératifs de création de logements, de responsabilité environnementale, de durabilité et de modularité de l'habitat. C'est pourquoi nous insistons

Ces élus de terrain, responsables au quotidien devant leurs électeurs, en ont un peu assez d'être dépossédés des attributions de logements au bénéfice de l'État ou des intercommunalités et de ne plus pouvoir répondre aux attentes des demandeurs locaux de logements. Ils en ont assez de cette marche forcée vers une forme de paupérisation de leur territoire, en particulier Comment voulez-vous, d'ailleurs, que les maires aient une appétence pour la construction de logements sociaux, si c'est pour y loger des populations qu'ils ne sont pas en mesure de gérer par la suite, tant elles posent de problèmes,

fixe le principe selon lequel « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir Cet amendement vise les personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de leur handicap, de leur grand âge ou en tant que personnes isolées,

de suivre et d'ajuster sa consommation de chauffage à partir des informations sur sa consommation réelle disponibles sur sa facture. Ce système limite les gaspillages en incitant les locataires à baisser la température. Le projet de loi prévoit que l'individualisation des frais de chauffage sera restreinte aux cas où le coût ne sera pas excessif et restera inférieur aux bénéfices attendus. Seulement, le texte actuel ne précise pas de quel coût il est question. Dans le cas d'une location, si l'on fait référence au coût pour le propriétaire, celui-ci peut n'avoir aucun intérêt à agir, les bénéfices attendus consistant en une diminution des coûts de chauffage pour le locataire. Il convient donc de préciser,

Le développement de l'autoconsommation d'électricité collective est devenu une priorité. Il doit être facilité, afin de répondre aux enjeux de la transition énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique. En effet, l'autoconsommation d'électricité contribue à développer la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et permet de maîtriser, voire de réduire, les factures d'énergie des ménages. Les organismes d'HLM se sont fortement engagés dans la mise en oeuvre d'opérations d'autoconsommation collective, en liaison avec

des échanges d'énergie entre plusieurs bâtiments, à finalités éventuellement différentes, dans le résidentiel ou dans le tertiaire. Il nous a semblé nous a semblé qu'il ne serait pas prudent d'aller au-delà, en particulier parce que les effets de l'autoconsommation collective sur les réseaux sont encore largement méconnus. J'ajoute que le législateur, en renvoyant à un arrêté, comme il est proposé, renoncerait à tout

l'acquisition de logements avec amélioration ou des travaux d'amélioration de logements existants, soit examinée la possibilité de mener des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des logements concernés. Les bénéficiaires des aides ne seraient évidemment pas contraints de réaliser ces travaux d'amélioration, mais ils seraient ainsi mieux sensibilisés à leur intérêt et incités à les réaliser concomitamment à d'autres travaux.

l'acte de construire sur nos territoires se confronte à des contraintes encore plus fortes et plus multiples qu'en France hexagonale. C'est une réalité. À ces nombreuses contraintes vient s'ajouter le poids de normes fréquemment en décalage avec les réalités ultramarines, ce qui conduit parfois à des situations ubuesques. Dans le cadre de son étude pluriannuelle sur l'impact des normes, la délégation sénatoriale aux outre-mer est remontée à l'origine du problème : « Les territoires ultramarins ne sont pas intégrés à la chaîne d'élaboration des normes réglementaires comme professionnelles. » Cela les laisse toujours dans l'angle mort, sans que leurs spécificités soient prises en compte. Aujourd'hui, force est de constater que la production des normes est répartie au sein du triangle formé par les services centraux du ministère, le Bureau de normalisation des techniques et équipements de la construction du bâtiment, le BNTEC, et le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, trois instances décisionnelles nationales desquelles les professionnels ultramarins peinent à se faire entendre et reconnaître. Par cet amendement, nous proposons donc d'assurer une représentation des départements et collectivités d'outre-mer dans le conseil d'administration du CSTB. En effet, ce dernier joue un rôle essentiel dans l'élaboration des réglementations et des normes, notamment par le biais de la Commission chargée de formuler les avis techniques, la CCFAT, dont il est membre et dont il anime les réunions d'experts. Il faut le dire, le poids de l'appréciation de la CCFAT est considérable et entraîne, en aval, le jugement des bureaux de contrôle et des assureurs, d'où l'importance d'y faire entendre la voix des outre-mer et de mieux prendre en compte leurs spécificités, pour pouvoir construire mieux et plus simplement. Quel

que le CSTB, dans le cadre de ses missions, accompagne la filière du bâtiment dans les transitions environnementale et numérique. Or l'État, ses opérateurs, les collectivités territoriales oeuvrent également pour cette mission d'intérêt général au travers de leurs politiques publiques et actions en matière de construction, d'habitat et de ville durable. Il convient donc, dans un souci de parallélisme, de mentionner que le CSTB leur apporte son concours.

Les climats particulièrement corrosifs et l'exposition accentuée aux risques naturels de ces territoires sont aujourd'hui insuffisamment pris en considération par le CSTB et la CCFAT. Il devient donc urgent de réviser la procédure d'avis technique, de manière que celle-ci intègre dorénavant la dimension ultramarine. À cet égard, plusieurs pistes ont été esquissées par la délégation aux outre-mer du Sénat adapter les avis techniques déjà délivrés au contexte ultramarin, permettre la délivrance d'avis techniques valables uniquement pour les outre-mer sur les produits innovants destinés à un usage en milieu tropical, rendre obligatoire la couverture des contextes ultramarins pour toutes les nouvelles demandes d'avis techniques, ou encore installer dans les outre-mer des relais régionaux du CSTB afin d'accompagner les entreprises ultramarines dans leurs démarches. Pour ce faire, nous proposons que la loi précise les missions du CSTB de manière à prendre véritablement en compte les spécificités ultramarines dans la procédure d'avis technique.

sera défavorable. Vous proposez en effet que le CSTB prenne en compte les spécificités, notamment climatiques, des départements d'outre-mer. Or, dans les travaux qu'il conduit, le CSTB

Or ils trouvent très peu de débouchés, alors qu'un chercheur qui travaille sur les normes environnementales dans l'Hexagone a des opportunités. Il faut donc que

La commission ne voit pas d'objection à préciser les dispositions législatives relatives aux modalités de contrôle du raccordement au service public d'assainissement.

pour les communes, qui devraient établir un diagnostic de conformité et réaliser des examens préalables avant travaux. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Merci